Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les finances locales sont au coeur de ce projet de loi de finances, et je tiens à revenir quelques instants L'article 5, que nous avons examiné en première partie, porte sur un sujet qui était très attendu : la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la réforme du financement des collectivités territoriales.

le Sénat. Ce décalage d'un an est sans incidence sur le contribuable, puisqu'il ne remet en cause ni la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2023 ni le dégrèvement total en faveur des 80 % des ménages les moins favorisés en 2020. Que le Gouvernement ne vienne pas nous dire que ce décalage n'est pas acceptable ou, pis, que c'est une mesure dilatoire : dans le même temps, il propose de ne réviser les valeurs locatives des locaux d'habitation qu'en 2026 Quand on sait l'importance de la distorsion de richesses imposée par la non-actualisation des valeurs locatives, on ne peut que déplorer ce calendrier. Ce décalage d'un an nous permettrait également de disposer du temps d'analyse et de concertation nécessaire pour traiter la question de la péréquation. Ce travail ne doit ne doit pas être mené à la va-vite, car il est vital, et pour cause : le reste de l'édifice financier local n'a plus de base tangible. La fiscalité est régulièrement réformée, souvent sans que les élus locaux le demandent ; les dotations sont dépassées, mais leur réforme n'est visiblement pas pour demain

Les autorisations d'engagement diminuent de 82 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2019. Toutefois, le montant des principales dotations en faveur du bloc communal demeure stable. Il représente, au total, 1,76 milliard d'euros en autorisations d'engagement. Au titre des crédits de paiement, la mission connaît une légère hausse pour 2020, de l'ordre de 13 millions d'euros. Ce solde masque néanmoins des mouvements parfois importants.

5 millions d'euros est versée à 1 122 communes dont une partie du territoire est couverte par une zone Natura 2000. Cette année, une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité est créée. Elle inclut l'ancienne dotation Natura 2000

voit transiter le produit des impositions locales versées mensuellement par l'État aux collectivités territoriales, qui devrait s'élever à 110,6 milliards d'euros en 2020. Nous vous proposerons d'adopter les crédits de cette mission et de ce compte de concours financiers. La parole

la mise en oeuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, sans toucher au bénéfice de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et en amendant le texte pour améliorer la compensation en faveur des collectivités.

C'est dans ce contexte que nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les articles qui y sont rattachés. Ce débat nous permettra de revenir sur un certain nombre de mauvaises manières faites aux collectivités territoriales- j'en évoquerai quelques-unes.

Il procède notamment à la réforme de la péréquation versée aux communes des départements d'outre-mer. Bien sûr, je salue cette mesure attendue depuis longtemps. Mais, une nouvelle fois, fort de son engagement envers les communes d'outre-mer, le Gouvernement laisse les autres communes financer cette réforme.

ne croyez pas que je veuille entrer maintenant dans des considérations techniques. Je relève simplement que cette décision du Gouvernement est révélatrice. Nous avions proposé ce report l'année dernière : il avait été balayé d'un revers de main. Finalement, le Gouvernement le reprend à son compte cette année. Nous en sommes heureux

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette année, la commission des lois n'a pas jugé utile de s'opposer à l'adoption des crédits ouverts au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »,

alors que nous nous sommes déjà prononcés sur une réforme de la fiscalité locale jugée, de l'avis général, prématurée, la commission des lois a souhaité attirer l'attention sur l'absence de prévisibilité des impacts d'une telle réforme sur les indicateurs financiers. Certes, ces impacts seront progressivement connus. Mais comment se fait-il qu'ils ne soient évalués qu'Plus généralement, la litanie des réformes de la fiscalité locale ne laisse pas aux collectivités territoriales le temps de s'adapter aux changements exigés d'elles. Ce qui est vrai pour la fiscalité l'est aussi pour les dotations d'investissement ou de fonctionnement que l'État attribue aux collectivités. Les élus ne sont ni convenablement informés ni suffisamment associés à des décisions d'attribution qui peuvent avoir un impact déterminant pour leur territoire.

L'attribution d'une part significative de cette dotation au niveau départemental et la création d'une commission départementale des investissements locaux, chargée de rendre des avis sur les décisions de subventionnement, permettraient de rapprocher les choix des besoins réels du terrain. créer une commission de suivi des investissements locaux chargée d'établir, en lien avec les services de l'État, la stratégie régionale de soutien de l'État à l'investissement local. La commission La commission des lois entend également s'opposer à la tentation recentralisatrice qui se fait souvent jour dans les modalités de répartition des dotations. L'an dernier déjà, elle s'est attachée à le démontrer : les vingt dernières années ont abouti à une recentralisation méthodique dans l'attribution des dotations d'investissement. Enfin, la commission des lois a souhaité apporter une solution à un problème récurrent : elle a voté un amendement important ayant pour objet le coefficient d'intégration fiscale et la dotation d'intercommunalité, dont les modalités de répartition ont une incidence directe sur l'organisation institutionnelle du bloc communal. À l'issue de l'examen de la mission RCT,

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

il est donc indispensable de prévoir en parallèle une remise à plat des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Chiche ! C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'un projet de loi de finances spécifique aux collectivités locales devrait être examiné par le Parlement chaque année. En second lieu, la préconisation du Sénat- reporter d'un an l'entrée en vigueur de la réforme -permettrait de solidifier le dispositif et d'éclaircir les zones d'ombre. Il faut bien le reconnaître : les élus ne sont pas rassurés, qu'il s'agisse du calcul du potentiel financier et fiscal ou de la compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation. Gardons en tête les atermoiements qui ont suivi certaines réformes mal préparées et leurs conséquences sur les collectivités. Nous ne voulons pas voir l'histoire se répéter

Au titre de la péréquation horizontale, la montée en puissance du FPIC ne permet pas réellement d'aplanir les écarts de richesse entre collectivités. Or les défauts de cet instrument sont de plus en plus manifestes. nous proposons plusieurs amendements : dans l'attente d'une réforme plus structurelle de révision des critères du FPIC, ces dispositions permettront pour le moins de ne pas trop pénaliser certains territoires qui bénéficient de la compensation de la taxe professionnelle. pour 2020 engage un alignement bienvenu des montants de péréquation alloués aux communes des départements d'outre-mer par rapport à la métropole. En outre, il amorce une réforme des modalités de répartition de cette enveloppe : nous l'approuvons, car elle renforce la solidarité nationale envers les communes d'outre-mer les plus pauvres et assumant le plus de charges. nous prenons acte de la traduction anticipée dans ce texte des mesures votées dans le cadre du projet de loi Engagement et proximité, conduisant à une majoration de la dotation particulière « élu local

Plusieurs amendements, dont certains déposés au nom du RDSE, visent justement à en modifier les modalités d'attribution afin de les rendre plus transparentes : je pense notamment à la commission DETR. Il faut saluer l'initiative du Gouvernement de pérenniser le soutien aux communes nouvelles dans un cadre clarifié pour les fusions qui suivront les élections municipales. De même, nous sommes favorables à la pérennisation du mécanisme de réalimentation des EPCI ayant une faible dotation.

a également été écartée., il faudrait exclure le surcroît de dépenses obligatoires induit par l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire du calcul de l'objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales.

Il faut bien le reconnaître : le Président de la République et le Gouvernement ont tenu leurs engagements en mettant fin à la baisse continue que les concours financiers de l'État aux collectivités locales subissaient

À cet égard, je souscris à la volonté de la commission des lois d'exiger davantage de transparence dans l'attribution des dotations ... Merci, cher collègue ! ... et une meilleure information des élus locaux. C'est pourquoi j'approuve les amendements adoptés, tendant notamment à créer une commission départementale des investissements locaux associant les élus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

de supprimer des formalités administratives et d'accélérer le versement des fonds aux collectivités locales. S'il est nécessaire d'approfondir l'évaluation financière d'une telle réforme, il serait incompréhensible,

du présent texte, les communes nouvelles percevront, au cours des trois années suivant leur création, une dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes. Le Gouvernement a donc respecté son engagement en introduisant de la souplesse et en maintenant l'enveloppe de la DGF dédiée au bloc communal à 27 milliards

S'agissant des flux financiers entre l'État et les collectivités territoriales et de leur rôle national en matière financière, économique et d'emploi, il en va un peu de

Ce qui devrait être le temps fort de la vie parlementaire, c'est-à-dire l'examen et le vote du projet de loi de finances, est devenu un théâtre d'ombres, un grand jeu de bonneteau destiné à masquer l'immobilisme politique de ces quinze dernières années. Avec le mois d'octobre revient le même pensum dont on connaît l'issue. On a beau répéter que la grille de lecture proposée ne permet pas de comprendre les enjeux, qu'intituler « Relations avec les collectivités territoriales » une mission budgétaire représentant 3,3 % seulement des transferts financiers de l'État ou 7,7 % des concours financiers auxdites collectivités est un non-sens, rien ne change. Plus que jamais, les choses absurdes doivent être faites dans les règles, sous peine d'apparaître pour ce qu'elles sont : absurdes. On félicitera donc nos rapporteurs d'avoir éclairé quelques ombres de ce trompe-l'oeil.

moins riches. De même, le « R » de cette même DETR n'est pas toujours visible dans tous les départements, d'où la proposition, bienvenue, de réserver une part de la dotation aux petites opérations. Ensuite, le mode de calcul du FPIC, censé évaluer la richesse des communes au sein des intercommunalités, est toujours aussi inique, puisqu'il favorise outrageusement les plus grandes d'entre elles en augmentant artificiellement leur population.

simple jeu de l'inflation et de la non-revalorisation des bases fiscales équivaudra à une charge supplémentaire de l'ordre de 2 milliards d'euros pour le budget des collectivités territoriales. Dans la novlangue budgétaire, les transferts financiers vont seulement de l'État vers les collectivités, et jamais dans l'autre sens. Ainsi sont présentés comme des « transferts financiers de l'État aux collectivités », donc comme des aides

pénalisant les collectivités, comme ce fut le cas avec la taxe professionnelle et comme ce le sera avec la taxe d'habitation, de captations d'impôts locaux particulièrement dynamiques,

la contrepartie, âprement discutée, de services rendus, le dernier en date étant les titres sécurisés, et bien d'autres décisions du même acabit. Parmi les curiosités les plus intéressantes, relevons le fait que les indemnités d'élus- dont les fonctions sont gratuites -payées par les collectivités, viennent, par le biais de l'impôt sur le revenu, abonder les recettes de l'État, ou encore que les dépenses de sécurité civile, une compétence de l'État exercée par les ministères de l'intérieur et de la santé, soient très largement

qui ne sont pas des compensations, sont plus proches de 35 milliards d'euros que des 115 milliards d'euros annoncés, lesquels ne tiennent évidemment pas compte des curiosités que je viens d'évoquer. Si j'ai tort, je ne demande qu'à être démenti par une étude exhaustive des flux financiers réels montants comme descendants entre l'État et les collectivités, étude qui, à ma connaissance, n'existe toujours pas.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » s'élèvent à 3,81 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 3,45 milliards d'euros en crédits de paiement pour 2020. Par rapport à l'année dernière, ils connaissent une baisse nette de 2,1 % en autorisations d'engagement tandis qu'ils augmentent légèrement, de 0,4 %, en crédits de paiement. Cette année encore, ils semblent témoigner d'une certaine défiance vis-à-vis des élus locaux, alors même qu'il faudrait, à l'évidence, essayer de rétablir la confiance Les dépenses des collectivités territoriales ont connu, depuis 2014, une très forte contrainte de la part de l'État. La baisse de 10 milliards d'euros, entre 2014 et 2017, des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales répondait ainsi à la volonté de voir ces dernières diminuer leurs dépenses d'autant.

son paroxysme au cours de l'actuel quinquennat - avec les contrats de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement, instaurés par la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, prévoit un dispositif de contractualisation destiné à maîtriser les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales. Or celles-ci sont les seules à respecter les contraintes budgétaires

On entretient à tort l'idée que les maires seraient de mauvais gestionnaires, on les prive de leur autonomie et ils ont parfois le sentiment d'être infantilisés. Pour ma part, je fais confiance aux élus locaux qui ont tracé des trajectoires vertueuses en réduisant leurs dépenses de fonctionnement pour se ménager des possibilités d'investissement. La réforme de la fiscalité locale prévue dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances, à l'article 5, va engendrer un nouveau bouleversement auquel les collectivités territoriales devront faire face et s'adapter.

destiné à neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la TFPB départementale aux communes. Les élus locaux sont ainsi confrontés à plusieurs incertitudes. En premier lieu, leurs inquiétudes concernent la perte, par les départements, d'une ressource sur laquelle ils bénéficiaient d'un pouvoir de taux. Madame la ministre, vous m'avez en partie répondu le 13 novembre

En second lieu, leurs préoccupations portent sur la réalité de la compensation « à l'euro près », promise par le Gouvernement, sur laquelle il est permis d'émettre des doutes eu égard aux expériences passées. C'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui amenés à examiner cette mission budgétaire. Aussi, je veux ici rendre un hommage appuyé à tous les maires des petites communes rurales, ces élus exemplaires qui ne comptent pas leur temps pour rendre service à leurs administrés, qui s'engagent au quotidien pour dynamiser leur territoire, pour créer du lien, avec bien souvent peu de moyens. Je veux saluer leur engagement au service de l'intérêt général.

territoriales », qui ne représente en réalité que 3 % des transferts financiers concernant les collectivités territoriales, offre des éléments de satisfaction. J'en citerai deux

Aussi, je salue la prise en compte de cette évolution législative permettant de maintenir une dotation forfaitaire qui « ne pourrait être inférieure à la somme des dotations perçues par chaque ancienne commune » l'année précédant la fusion.

plus de transparence et permettra aux élus nationaux d'être davantage partie prenante dans l'attribution de ces crédits. S'agissant des dotations de compensation,

proviendrait d'un transfert de dotations en provenance des départements et des régions. Cela nous laisse perplexes : nous remercions les départements et les régions, lesquels, à l'insu de leur plein gré, seront ainsi amenés

à garantir la neutralisation financière des restitutions de compétences par les EPCI à leurs communes membres, une disposition que nous avions défendue, avec mon collègue corapporteur Mathieu Darnaud, lors de l'examen du projet de loi Engagement et proximité, et qui a déjà été présentée

Cette mission « Relations avec les collectivités territoriales » s'inscrit dans un contexte singulier plus large. Je ne peux pas ne pas évoquer la réforme de la taxe d'habitation, qui représente 36 % des ressources des communes et des EPCI. Certes, je reconnais bien volontiers que cet impôt est très inéquitable.

heurte le principe d'autonomie fiscale et financière des collectivités et leur sens des responsabilités, même si je reconnais qu'il y a là un effet péréquateur pour les départements qui n'existait pas au préalable : c'est un bienfait.

Les subventions d'investissement aux collectivités territoriales sont reconduites en 2020, à hauteur de 2 milliards d'euros, avec notamment 1 milliard d'euros affectés à la dotation d'équipement aux territoires ruraux (DETR), chère à nos maires. Par ailleurs, la dotation de solidarité rurale (DSR) augmente en 2020 de 90 millions d'euros, comme en 2019. Les élus que je rencontre dans l'Eure- un territoire rural -se posent toutefois les questions suivantes. Tout d'abord, la suppression de la taxe d'habitation sera-t-elle compensée à l'euro près ? Ensuite, la hausse des dotations de péréquation verticale impliquera-t-elle la diminution d'autres dotations ? Enfin, cette péréquation, qui bénéficie aux territoires ruraux, sera-t-elle bouleversée dans les années à venir ? Les maires attendent en effet la réforme de la fiscalité locale prévue en 2021. S'agissant du premier motif d'inquiétude, le projet de loi Engagement et proximité prévoit que la fraction de la taxe d'habitation perçue par le département soit versée en compensation de celle que perdent les communes. Ce système semble judicieux et nous espérons qu'il fonctionnera dès l'an prochain. Sur le deuxième motif d'inquiétude, je rappelle que la hausse de 190 millions d'euros de la péréquation verticale est financée par les collectivités locales elles-mêmes, au travers d'écrêtements qui entraînent des baisses de dotation forfaitaire pour de nombreuses communes rurales. cela s'ajoute une minoration des variables d'ajustement à hauteur de 122 millions d'euros. Pour respecter les plafonds fixés par l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, l'État doit en effet compenser toute hausse en diminuant d'autres dotations.

départementaux de péréquation de cette même taxe, et enfin à la totalité de la dotation compensant les transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale. En 2018, l'assiette a intégré la DCRTP du bloc communal en 2020, elle sera étendue au prélèvement sur recettes (PSR) qui compense les exonérations relatives au versement transport. Toutefois, certaines mesures techniques ont été prises en sens inverse. Ainsi, la dotation sera réduite à 75 millions d'euros en 2020, dont 10 millions d'euros en moins pour le bloc communal, ce qui constitue un sujet d'inquiétude pour les élus. Le relèvement du seuil de neuf à onze salariés pour les entreprises a diminué de moitié la compensation du versement transport. Cela ne va pas encourager le développement du transport collectif, indispensable dans nos territoires ruraux. Par ailleurs, les élus de nos territoires ruraux s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir la réforme de la fiscalité locale sur les montants de péréquation. La suppression des bases de salaires de la taxe professionnelle (TP) en 2005, la disparition définitive de la TP en 2012 ou encore les fusions opérées par la loi NOTRe en 2018 ont entraîné des modifications fiscales profondes. La péréquation horizontale, mais aussi verticale, sera impactée en 2020 : le critère du potentiel fiscal par habitant est utilisé dans six mécanismes et constitue l'une des

En effet, ces territoires vont voir leur potentiel financier augmenter par rapport à la moyenne nationale, et donc percevoir moins de péréquation. Madame la ministre, si l'on peut se satisfaire de certaines décisions prises en faveur des collectivités territoriales, il serait souhaitable que des simulations soient portées à la connaissance des parlementaires pour éclairer leur jugement et rassurer les élus de nos territoires. Madame la ministre, il faut écouter le Sénat ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est difficile de réduire l'examen des relations entre l'État et les collectivités à l'analyse de la seule mission qui nous réunit aujourd'hui, d'un montant de 3,8 milliards d'euros, quand l'ensemble des concours financiers s'élèvent à 48,9 milliards d'euros et que la principale nouveauté pour les collectivités se trouve à l'article 5 de ce projet de loi de finances et concerne la suppression de la taxe d'habitation.

À y regarder de plus près, je crains, malheureusement, qu'elle ne fasse surtout beaucoup de perdants, d'abord, parmi les contribuables. Si 29,5 millions de foyers sont assujettis à la taxe d'habitation, 5,1 millions ne la paient pas. Pour eux, les plus modestes, le gain de pouvoir d'achat est égal à zéro. Pour les 80 % qui en bénéficient déjà, le gain moyen sera de 555 euros en 2020. Pour les 20 % restants, les plus aisés, le gain sera de 1 158 euros en 2023 même, si l'on en croit notre estimé collègue M. Alain Richard, 2 035 euros pour les foyers relevant de la tranche à 45 % de l'impôt sur le revenu. En résumé : quand vous êtes pauvre, vous ne gagnez rien ; plus vous êtes riches, plus vous gagnez À l'inégalité sociale s'ajoute une égalité territoriale, car supprimer la taxe d'habitation avant d'engager la révision des valeurs locatives, repoussée aux calendes grecques, revient à fossiliser les différences de situation. Les communes qui avaient un produit inférieur à la moyenne, en raison d'une assiette réduite souvent liée à une population modeste, recevront une compensation inférieure à la moyenne, sans espoir de rattrapage. Les communes pauvres seront donc perdantes. Ainsi, annoncer la suppression d'un impôt injuste ne revient pas à oeuvrer pour la justice fiscale

d'une part parce que la compensation se fera sur la base des taux de 2017, gommant les augmentations de ces deux dernières années démocratiquement décidées par des municipalités souvent contraintes par des difficultés financières. Cela représente une perte de recettes supérieure à 100 millions d'euros, que le Gouvernement n'hésitera d'ailleurs pas à empocher. D'autre part, après avoir envisagé de déroger à la revalorisation forfaitaire obligatoire des valeurs locatives, qui aurait provoqué un manque à gagner de 250 millions d'euros, le Gouvernement s'est rangé à la position de l'Assemblée nationale qui a corrigé le tir en se limitant toutefois à une augmentation de 0,9 %, inférieure au chiffre de 1,2 % de l'indice des prix à la consommation harmonisé. La perte de recettes atteindra donc 140 millions d'euros. Tous seront perdants, toujours, sur les dotations. Cette réforme aura des conséquences considérables sur le potentiel financier, lequel pourrait varier dans des proportions d'un tiers, à la baisse ou à la hausse, par rapport à la moyenne nationale. Personne aujourd'hui ne dispose de simulation des conséquences possibles sur la vingtaine de dotations qui seront concernées. Des pauvres deviendraient subitement riches et seraient privés de soutien, quand des riches y deviendraient éligibles C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu la proposition du rapporteur général de la commission des finances de reporter d'un an la mise en oeuvre de la compensation et de maintenir le dégrèvement avant d'y voir plus clair. Perdants, enfin, les départements, qui voient un impôt dynamique disparaître. Le transfert de la part de foncier bâti compensé par l'attribution d'une fraction de TVA à compter de 2021 affaiblira l'évolution de leurs recettes fiscales, puisque, entre 2005 et 2017, le dynamisme de la TVA, de 2,07 % par an, était inférieur à celui de l'évolution des bases de foncier bâti, lesquelles ont progressé dans la même période de 3,13 %. Si la réforme avait été appliquée depuis 2005, les départements auraient ainsi perdu 4 milliards d'euros de recettes. Autrement dit, ils récupèrent une recette fiscale sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir de taux et qui pourra baisser d'une année sur l'autre. Madame la ministre, cette réforme bouscule et déstabilise la structure des recettes de nos collectivités territoriales ; elle rompt le lien entre le citoyen et le territoire et attaque le consentement à l'impôt elle supprime le dernier impôt local universel du bloc communal, gèle le pouvoir de taux de celui-ci et annule presque totalement l'autonomie fiscale des départements. Bref, elle est contraire à l'esprit de la décentralisation

vous avez bénéficié d'une situation assainie, avec un déficit ramené sous la barre des 3 % et une croissance retrouvée qui vous offrait des marges de manoeuvre, dont vous n'avez à aucun moment fait profiter les collectivités

Rien dans ces 600 millions d'euros ne correspond à une décision nouvelle ; il ne s'agit que d'obligations légales. Ainsi, 350 millions d'euros proviennent du dynamisme du FCTVA, qui progresse parce que l'investissement des collectivités territoriales 128 millions d'euros correspondent à la fraction de TVA accordée aux régions en remplacement de la DGF, car la TVA cette année est dynamique. Enfin, 123 millions d'euros sont liés à la progression des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale votées les années précédentes,

vous intégrez un nouveau concours financier au périmètre des variables d'ajustement, pour compenser aux collectivités territoriales les pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. Cette compensation dynamique, d'un montant de 93 millions d'euros pour l'année à venir, est désormais plafonnée à 48 millions d'euros, ce qui entraîne une baisse de 45 millions d'euros une compensation de plus qui, censée couvrir intégralement des pertes de recettes- ici, pour les autorités organisatrices de transport -, n'est pas complète. Pour la première fois, la minoration des variables d'ajustement servira aussi à gager une mesure qui n'entre pas dans les concours financiers de l'État aux collectivités

Son principal dispositif, le FPIC, qui a fortement participé à la réduction des inégalités, à hauteur de 1 milliard d'euros, est malheureusement encore gelé, alors que les recettes fiscales des communes les plus riches continuent de progresser. La péréquation verticale, par définition, devrait être assurée par l'État. Pourtant, depuis 2018, vous la détournez en gageant son augmentation au sein de la DGF sur la baisse de la dotation forfaitaire.

De même, la réforme de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, qui assure un rattrapage bienvenu de 17 millions d'euros par rapport aux communes de l'Hexagone, sera financée sur des minorations au sein de la DGF plutôt que par de l'argent frais. Ajoutons à cela que certaines communes riches, ayant une DGF nulle, ne contribuent pas à la péréquation. L'ensemble de ce dispositif explique que, l'année prochaine encore, plus de la moitié des communes verront leur DGF baisser, l'État leur faisant payer le coût de ses engagements finances marque un ralentissement du soutien à l'investissement local. Sous le précédent quinquennat, les dotations de soutien à l'investissement avaient fortement progressé, pour conforter ce moteur de croissance qui représente plus de 70 % de l'investissement public civil.

: loin de traduire un soutien massif de l'État aux collectivités territoriales, ce projet de loi de finances fragilise leurs moyens financiers en réduisant insidieusement leurs dotations et en affaiblissant brutalement leur pouvoir fiscal.

Nous pourrions accueillir cette nouvelle avec satisfaction- si la réalité n'était pas tout autre ... Sur le papier, à la lecture des articles rattachés aux crédits de cette mission, les moyens alloués à la dotation globale de fonctionnement sont stables ; dans les faits, toutefois, ils se dégradent. En effet, comme l'an dernier, ils ne prennent en compte ni l'augmentation de la population dans les communes ni l'inflation : en euros constants, nous sommes bien face à une diminution. Malgré les multiples opérations de séduction du Gouvernement, les élus locaux ne sont pas dupes ! Derrière les discours, vous ne leur accordez pas l'essentiel, le pendant de leur liberté d'agir : les moyens de leur autonomie financière et fiscale, pourtant consacrée par notre Constitution et par de nombreux textes européens auxquels nous sommes attachés. La libre administration, c'est-à-dire la responsabilité des politiques que les élus locaux mènent sur leur territoire, est indissociable de la responsabilité fiscale et budgétaire, donc de l'autonomie des collectivités territoriales.

affiché des finances publiques et réduit la voilure- là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. pour 2020 enfonce le clou un peu plus, avec la suppression de la taxe d'habitation à l'horizon de 2023. Encore une fois, l'État choisit de supprimer un impôt qui ne lui appartient pas

il convient de ne pas les fragiliser ! Aujourd'hui, nous sommes bien loin de la promesse faite par le Gouvernement de compenser à l'euro près le dégrèvement de la taxe d'habitation. Deux ans après les annonces, nous découvrons que la compensation se fondera sur des règles que nous n'aurions jamais imaginées

Certains territoires que je connais bien subissent souvent une double peine fiscale. D'abord, les DGF dites négatives posent de vraies difficultés pratiques. C'est vrai ! La contribution au redressement des finances publiques est prélevée sur la DGF ; quand celle-ci n'est pas suffisante, le solde manquant est ponctionné sur les recettes fiscales.

Ces deux phénomènes obèrent de façon très importante les capacités financières des communes concernées, qui doivent pourtant assumer des investissements spécifiques et lourds liés à leurs caractéristiques frontalières et montagnardes. Il ne s'agit nullement de remettre en cause les principes de péréquation et de solidarité, mais de cesser de faire peser sur ces territoires une part déraisonnable et disproportionnée de la péréquation horizontale.

il implique, au minimum, qu'elles entretiennent des liens fondés sur la confiance. La question centrale est donc simple : cette mission budgétaire garantit-elle la confiance entre l'État et les collectivités territoriales ? Avant d'y répondre, il convient de remettre la question en perspective.

principe « faire mieux avec moins » a atteint ses limites. Pourtant, personne ici ne peut remettre en cause ce fait simple : c'est aux collectivités territoriales, non à l'État, que nous devons la plus grande contribution à la réduction du déficit public.

En 2020, une fois encore, l'effort de maîtrise de la dépense publique reposera surtout sur les administrations publiques locales- à 31 %, contre 22 % pour l'État et ses opérateurs.

Certes, les niveaux de la DETR et de la dotation de soutien à l'investissement sont maintenus, mais nous n'avons pas oublié, et les maires non plus, la disparition de la réserve parlementaire, sacrifiée à l'air du temps et confiée pour partie seulement aux préfets : un exemple de plus du manque de confiance

Ainsi, en mars prochain, au lendemain des élections municipales, les nouveaux élus ne pourront pas délibérer sur le taux de taxe d'habitation. En outre, le Gouvernement envisage d'annuler en 2020 les effets des augmentations de taux décidées par les communes et les EPCI en 2018 et en 2019. Pour la taxe d'habitation sur les locaux vacants, ce gel des effets des délibérations perdurera même jusqu'en 2023 ! Au total, ce dispositif conduit à une perte de recettes de 160 millions d'euros pour les collectivités De plus, le Gouvernement semble s'opposer à toute revalorisation forfaitaire des bases en 2020. Cette mesure réduira aussi les ressources locales, de 250 millions d'euros par an environ.

la non-indexation de ces dotations sur l'inflation et l'absence de prise en compte de l'augmentation de la population, soit une perte sèche de 600 millions d'euros par an pour la seule DGF.

... À tort ou à raison, nombre d'élus ont le sentiment que la politique de contrôle, parfois tatillon, de réduction des moyens et de recentralisation se poursuit, et que les liens continuent à se distendre entre le centre et les territoires. Aussi, comme nombre de mes collègues, j'attends avec impatience le projet de loi « décentralisation, déconcentration déconcentration et différenciation » que vous êtes appelée à défendre, madame la ministre. Puisse-t-il ne pas être un nouveau rendez-vous manqué ... Le Sénat sera au rendez-vous, le Gouvernement doit l'être aussi ! Sous réserve de l'adoption de certains amendements, issus en particulier de la commission des lois, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission.

Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2017, le Gouvernement présente des budgets en rupture avec les pratiques antérieures et reposant sur trois piliers

Je ne reviendrai pas sur ces dispositions fiscales d'ampleur, dont le principe peut être résumé en une formule : 18 milliards d'euros de réduction d'impôts pour les Français et

qui visent les dépenses de fonctionnement des 322 collectivités territoriales aux budgets les plus importants. Ce dispositif a produit ses premiers résultats en 2018

mais les finances de notre pays sont ce qu'elles sont : on ne peut pas nous demander à la fois d'arrêter de creuser le déficit et de prendre des mesures qui le creuseraient

les députés ont voté une majoration de 20 millions d'euros, reprenant la progression des années précédentes, interrompue en 2019. S'agissant de la garantie de sortie du FPIC, elle a été unifiée et améliorée pour plus d'une centaine d'ensembles

car le Gouvernement a clairement annoncé que les indicateurs financiers des communes, des EPCI et des départements devraient être revus après la réforme fiscale, pour neutraliser les effets de bord

Lors du « printemps de l'évaluation », certains d'entre vous ont insisté sur la nécessité de mieux évaluer aussi l'impact de la péréquation. Ce travail d'évaluation pourra rejoindre,

Je veillerai à ce que le Parlement, en particulier les délégations aux collectivités territoriales, soit associé en amont à ce travail et aux simulations menées.

a déjà signalé celle qui concerne l'accompagnement financier de la création de communes nouvelles. Depuis 2015, le pacte de stabilité sur la DGF des communes nouvelles a facilité un nombre important de regroupements communaux. Néanmoins, les critères d'éligibilité aux avantages du pacte ont fait l'objet d'une certaine instabilité, ce qui ne permettait pas aux élus de préparer leur fusion

avec les mêmes seuils qu'aujourd'hui, de garanties sur le montant de leurs attributions au titre de la dotation forfaitaire, ainsi que de dotations de péréquation, pendant les trois années suivant leur création.

EPCI. Un certain nombre d'élus souhaitaient une plus grande responsabilité locale : nous avons entendu ce besoin de responsabilité et prévu une capacité d'agir localement sur la répartition de la DGF des communes. d'une possibilité. Le constat est simple : la DGF est répartie selon des critères nationaux, qui ne peuvent pas traduire l'ensemble des caractéristiques locales et des spécificités de chaque territoire.

DGF. À l'heure actuelle, les communes membres d'un même EPCI ne disposent pas d'un levier efficace pour opérer une répartition différente de la DGF, quand bien même elles seraient d'accord pour le faire. Nous proposons donc un système simple et- j'insiste -facultatif de répartition dérogatoire de la DGF des communes au sein d'un EPCI, sous réserve de l'accord de toutes les communes et selon les critères qu'elles estiment le plus adaptés à leurs caractéristiques.

Elle se traduit par certains engagements de compensation de mesures nouvelles, comme l'obligation de souscrire un contrat d'assurance de protection fonctionnelle ou le remboursement des frais de garde de jeunes enfants.

Au total, l'État engage 2 milliards d'euros en 2018, en 2019 et en 2020 au titre de la mission RCT pour soutenir l'investissement local. Les modalités de gestion de ces concours ont beaucoup évolué ces deux dernières années,

Le Président de la République a annoncé l'engagement d'une démarche de rattrapage financier de l'outre-mer sur cinq ans, entre 2020 et 2024. de finances est la première étape de ce rattrapage. Elle conduit à augmenter la péréquation dans les DOM de 19 millions d'euros entre 2019 et 2020, d'euros par rapport au droit en vigueur. Les communes des DOM bénéficient aujourd'hui de la péréquation verticale dans des conditions dérogatoires qui soulèvent deux difficultés les montants alloués sont inférieurs d'environ 55 millions d'euros à ceux qui résulteraient du droit commun et les critères de répartition ne permettent pas de cibler les communes les plus fragiles. Suivant les recommandations du Comité des finances locales, ce surcroît est réparti de manière péréquatrice pour aider les communes qui en ont le plus besoin. Cette majoration s'inscrit dans une démarche plus large visant à mieux assurer l'autonomie financière des communes d'outre-mer en agissant tant sur leurs recettes- DGF, meilleur recensement des bases fiscales-que sur la structure de leurs dépenses. La mission confiée par le Gouvernement au sénateur Georges Jean-René Cazeneuve doit proposer prochainement de nouveaux outils d'accompagnement et de contrôle. Je souhaite que, si c'est possible, notre réforme de la Dacom puisse tenir compte de leurs conclusions. Un autre sujet

de la péréquation horizontale entre départements, le Gouvernement a fait adopter par l'Assemblée nationale un amendement dont le dispositif- je tiens

Par ailleurs, à compter de 2021, un fonds de péréquation financé grâce à la dynamique

À la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement visant à créer une dotation de soutien aux communes pour la protection de l'environnement, il convient d'abonder le programme 119 à hauteur de 5 millions d'euros.

Je voterai cet amendement. Toutefois, le problème de fond reste entier et on refuse de l'examiner

Je persiste à penser que c'est un pur scandale

Cet amendement vise à porter les crédits de la dotation de soutien à l'investissement local à son niveau de 2018, à savoir 615 millions d'euros en autorisations d'engagement. Afin de respecter les exigences de l'article 40 de la Constitution, nous prévoyons une diminution de 45 millions d'euros

est ainsi libellé : La parole est à M. Yves Daudigny. Cet amendement vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses des communes liées à l'activité de domiciliation des personnes sans domicile par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale,

Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un grand nombre de démarches.

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », en réduisant d'autant les crédits de l'action n° 02, Administration des relations avec les collectivités territoriales, du programme 122 Ces crédits ont notamment pour objet de financer les dépenses d'investissement nécessaires afin d'augmenter les capacités d'accueil des services de domiciliation actuels des communes, réhabiliter des locaux ou acheter du matériel. Toutefois, la dotation générale de décentralisation, la DGD, est une ressource de la section de fonctionnement et ne peut donc financer directement de telles dépenses d'investissement, qui, par ailleurs, sont très variables selon les collectivités. En outre, la création d'une DGD spécifique ne nous semble pas appropriée. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

par les CCAS, ne constitue pas un transfert de compétences au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle ne nécessite donc pas de compensation.

concerne la sécurité de l'ensemble des Français. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Mirepoix-sur-Tarn ne résulte pas d'un défaut d'entretien- nous sommes bien d'accord -, mais cela a mis en lumière,

J'ai évoqué tout à l'heure la question du dédoublement des classes de CP. On pourrait aussi évoquer les besoins en matière d'accès à la culture et aux activités sportives, de soutien à la vie associative : ils nécessitent des investissements que bon nombre de ces communes

Une mobilisation de l'État est alors indispensable. Les dispositifs actuels, comme les subventions exceptionnelles de fonctionnement de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », ne sont pas dimensionnés pour répondre à ce besoin.

au soutien, dans le cadre de contrats d'accompagnement renouvelés, des collectivités pour lesquelles une aide extérieure est indispensable.

d'étudier votre proposition ... En outre, en minorant le programme 119, l'amendement tendrait à diminuer le montant des dotations d'investissement, ainsi que des dotations générales de décentralisation qui sont dues.

La Caraïbe, pour la partie qui me concerne le plus, fait en effet partie des zones les plus vulnérables et, pourtant, les moins productrices de gaz à effet de serre. Au quotidien, nos communes sont obligées d'affronter, avec responsabilité et courage,

et l'on continue de s'enfoncer, loin des plans de redressement qui pourraient venir ici ou là. Je plaide donc pour que les différences structurelles de financement de ces communes soient définitivement prises en compte. On nous annonce un grand soir pour l'année 2020

aussi des actes ! Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix ces crédits, modifiés.